La séance est reprise. Monsieur le Premier ministre, mesdames, messieurs les ministres, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle les réponses à des questions d'actualité au Gouvernement.

Je vous rappelle que la séance est retransmise en direct sur Public Sénat, sur le site internet du Sénat et sur Facebook. Au nom du bureau du Sénat, j'appelle chacun d'entre vous, mes chers collègues, à observer au cours de nos échanges l'une des valeurs essentielles du Sénat : le respect, qu'il s'agisse du respect des uns et des autres ou de celui du temps de parole. La parole est à M. Jean-Marie Bockel, pour le groupe Union Centriste. Union Centriste. En mai, puis le 13 juin dernier, des attaques ont eu lieu dans le détroit d'Ormuz, en mer d'Oman, symbolisant la montée des périls dans la région du Golfe depuis plusieurs mois. Nous avons tous à l'esprit les images de navires en flammes diffusées sur nos écrans. Sur fond de remise en cause du traité sur le nucléaire, les tensions s'exacerbent entre Washington et Téhéran, mais aussi entre leurs alliés respectifs. Déjà, on parle de risque de guerre. Les hostilités peuvent se déclencher à la moindre étincelle, presque par accident. L'attitude de la France est scrutée, du fait de sa capacité à parler avec tous les acteurs de la région et de son statut de membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Quelles nouvelles initiatives peut-elle prendre pour éviter le déclenchement d'un conflit dont les conséquences seraient tragiques ? J'ajoute que notre implication dans les enjeux du Golfe ne saurait se limiter à notre seul engagement diplomatique. Ainsi, la France a conclu, avec raison, des accords stratégiques avec plusieurs pays de la région, dont l'Arabie saoudite., ces accords, ces accords, notamment ceux qui portent sur les ventes d'armes, nous inscrivent dans le conflit au Yémen : une « sale guerre », comme le dit M. Le Drian. Nécessaires à la survie de notre industrie de défense, nos ventes d'armes respectent, selon vos dires, le traité sur le commerce des armes, notamment ses articles 6 et 7. J'ai à l'esprit la vigilance de plusieurs ministres sur les livraisons d'armes. Elles n'en font pas moins débat. À l'heure où se tient le salon du Bourget, qui fait notre fierté, y compris en matière d'armement, quelle est notre action en faveur du cessez-le-feu et de la sortie de ce conflit effroyable ? La parole

est dans l'intérêt de la sécurité de la France, de l'Europe et du monde. Cette conviction a guidé notre action tout au long de ces derniers mois, en dépit du retrait américain, intervenu voilà plus d'un an. Nous avons récemment assisté à une montée des tensions et des provocations dans les eaux du golfe Persique et au-delà. Les derniers incidents impliquant des pétroliers en mer d'Oman contribuent à alimenter des tensions déjà fortes ; toute la lumière doit être faite sur ces événements. Il importe d'éviter une escalade non maîtrisée et de privilégier le dialogue pour réduire les tensions. La priorité est que l'Iran reste partie à l'accord sur

L'Iran doit pouvoir bénéficier de l'accord de Vienne, comme celui-ci le prévoit. Toutes les parties doivent rechercher la voie d'une désescalade par des gestes discrets et modestes ; le Gouvernement travaille en ce sens. le second volet de votre question, le peuple yéménite subit effectivement une terrible crise humanitaire dans ce conflit qui n'a que trop duré. Les pourparlers qui se sont tenus en décembre en Suède, sous l'égide des Nations unies, ont permis, pour la première fois depuis des années, d'ouvrir une perspective de paix. Leurs résultats ont été endossés par le Conseil de sécurité. Une mission d'observation des Nations unies a été déployée sur le terrain dans la ville côtière d'Hodeïda. Les parties observent dans cette ville et alentour une trêve, qui est relativement bien respectée. La médiation des États-Unis au travers de l'action de l'envoyé spécial du secrétaire général, Martin Griffiths, cherche à obtenir un accord global rassemblant toutes les parties yéménites. La France s'emploie à faire aboutir ces efforts de paix, auprès tant du gouvernement yéménite que des Houthis

vignes, abricotiers, noyers, serres, toitures, voitures, écoles, bâtiments publics, monuments historiques, rien n'a été épargné. Une personne a même perdu la vie en Haute-Savoie, et le bilan aurait pu être bien plus lourd. Au vu de l'état de l'école primaire et maternelle de Châtillon-Saint-Jean, on comprend que le pire aurait pu survenir si ce phénomène s'était produit un jour scolaire. Vous avez vous-même pu le constater dimanche et lundi derniers. Je salue celles et ceux dont la mobilisation et l'engagement ont permis de limiter les conséquences de cette catastrophe : sapeurs-pompiers, policiers, gendarmes, personnel municipal, dont le courage et le professionnalisme ont permis une prise en charge très rapide des situations les plus graves. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir relayé directement auprès des services de secours le message de reconnaissance du Président de la République et d'être venu immédiatement au chevet de celles et de ceux qui ont tout perdu, de ceux que vous défendez sans relâche

Aujourd'hui, le temps est venu de panser les plaies, ce que vous avez commencé à faire en rassurant sur les procédures qui vont être mises en place. Reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, dispositif relatif aux calamités agricoles, exonération ou allégement de certaines charges à la suite des pertes d'exploitation, chômage des personnels agricoles : agriculteurs, particuliers

Le week-end dernier, cela vient d'être rappelé, la région Auvergne-Rhône-Alpes a été frappée par de violentes intempéries. Cette nuit, dans ma région, c'est la ville de Toulouse qui était en proie à des vents et des orages d'une force rare. Ces événements ont occasionné des dizaines de millions d'euros de dégâts et, une fois de plus, les agriculteurs se retrouvent en première ligne, parmi les plus sinistrés.

Dans ces conditions, l'avenir s'annonce encore bien sombre pour de nombreux agriculteurs, qui voient régulièrement l'investissement de toute une année ruiné en quelques minutes. Monsieur le ministre, vous avez rapidement annoncé la déclaration de l'état de catastrophe naturelle et la

contre la grêle. Par ailleurs, les dispositifs de protection, les filets sont trop coûteux et pas toujours efficaces. Au-delà des aides à court terme de l'État, ne faudrait-il pas surtout bâtir un système assurantiel

référendum sur la privatisation d'Aéroports de Paris est lancée. C'est une première, une expérience démocratique inédite, portant sur un enjeu d'intérêt national : il s'agit de savoir si la plus grande plateforme aéroportuaire de France, l'une des toutes premières au monde, restera publique ou sera livrée aux actionnaires, comme les autoroutes Or, du côté du Gouvernement, depuis une semaine, c'est le silence radio : une ouverture du site internet le 13 juin en catimini ; aucune allusion dans les deux déclarations de politique générale aucun compte rendu public de la rencontre organisée entre le ministre de l'intérieur et les parlementaires issus de toutes les familles politiques à l'initiative de cette démarche. Je comprends que vous ayez du mal à digérer l'affaire, mais il va falloir vous y faire : si le site officiel ne comporte pour le moment aucun compteur, une association spécialiste du numérique en a créé un, qui relevait déjà ce matin 235 832 signatures. Pourtant, au ministère, des annonces nous ont été faites, qui méritent d'être connues de tous : outre les personnes déjà inscrites sur les listes électorales, les nouveaux inscrits pourront participer ; plusieurs citoyens peuvent enregistrer leur signature à partir d'une même adresse IP ; toutes les communes peuvent devenir point d'accueil des signatures si elles se portent volontaires. Trois questions restent en suspens, monsieur le ministre : comment comptez-vous élargir la communication au grand public et allez-vous organiser une grande campagne d'information civique ?

Envisagez-vous une refonte globale de la plateforme, qui n'est absolument pas ergonomique par comparaison avec le site du grand débat ? Le comité de suivi va-t-il se mettre en place, et si Quand et selon quel rythme y aura-t-il une communication sur le nombre de signatures recueillies ? Les internautes ont prouvé la faisabilité technique d'un décompte au fil de l'eau. Monsieur le Premier ministre, le référendum d'initiative partagée est de valeur constitutionnelle. Il incombe au Gouvernement de le mettre en oeuvre dans les meilleures conditions possible. Ce n'est pas le cas pour l'instant.

Il y a ici un axe républicain, un arc républicain, pour demander de la transparence, tout simplement, conformément à l'esprit, monsieur le Premier ministre, de l'article 3 de la Constitution, dont je me permets de rappeler les termes : « La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. est à Mme Colette Mélot, pour le groupe Les Indépendants-République et Territoires.

le monde a besoin d'une devise numérique mondiale qui combine les attributs des meilleures devises du monde : elle doit être stable, soumise à une inflation faible, acceptée partout dans le monde et fongible c'est ainsi que Facebook présente une nouvelle monnaie destinée à payer des services en ligne, mais aussi son loyer ou son café. Croire à une démarche philanthropique serait oublier bien vite que toutes nos données sont conservées et utilisées par les géants du numérique pour, aujourd'hui, nous envoyer des publicités ciblées, et peut-être, demain, les utiliser à des fins moins

en Suisse, Calibra. Comment croire que les données financières seront bien séparées des données sociales, alors même que les fuites et les mauvais usages de données sont déjà récurrents ?

Comment être convaincu des bonnes intentions de ces grandes sociétés ? Les Gafam cachent à peine leurs ambitions : Google gérera bientôt une ville dans la métropole de Toronto et se propose de régler la crise du logement à San Francisco. Monsieur le ministre, cette nouvelle monnaie suscite de nombreuses inquiétudes, et vous avez déjà fait à son propos des déclarations qui se veulent rassurantes. Devant un risque de remise en cause de l'État, que comptez-vous faire pour anticiper au mieux ces évolutions et protéger les Français ? Ce combat sera-t-il mené au niveau européen ? La parole

Elle est libre de créer un instrument de transaction ; en revanche, elle ne peut pas et elle ne doit pas mettre en place une monnaie souveraine : seuls les États ont la capacité et la légitimité de le faire.

C'est sur la base des propositions des gouverneurs des banques centrales des États membres du G7 que nous prendrons les décisions nécessaires. Je rappelle enfin que cet instrument

du jamais vu » : c'est ce que les agriculteurs nous ont dit après avoir constaté les dégâts considérables provoqués par la grêle dans notre département. Ces dégâts ne concernent pas seulement la Drôme : je souhaite associer à cette question mes collègues de l'Ardèche, de l'Isère, de la Savoie et de la Haute-Savoie. Ces départements n'ont pas eu l'honneur de votre visite, mais ils ont également été durement touchés. C'est toute une économie qui est mise à mal. Les agriculteurs et les viticulteurs ont besoin de la solidarité nationale, faute de quoi ils mettront la clé sous la porte.

Monsieur le ministre, si l'État ne procède pas au cas par cas et n'accompagne pas plus largement les agriculteurs, nous assisterons à des faillites. Que comptez-vous faire de concret et d'efficace pour répondre à toutes les situations de détresse ?

L'avenir de l'alliance Renault-Nissan sera certainement au coeur des discussions. Dans ce contexte, on ne peut pas faire comme si de rien n'était quant au sort de notre compatriote Carlos Ghosn, ex-PDG du groupe, qui a redressé Renault, relocalisé l'emploi industriel en France, sauvé Nissan et Mitsubishi. Très bien ! Nous ne connaissons pas les accusations portées à son encontre et ne pouvons donc pas en mesurer la gravité et la pertinence. Par conséquent, aucun commentaire n'est possible sur le fond. Toutefois, le Japon agit en violation de ses propres engagements internationaux. Depuis plus de sept mois,

Par ailleurs, comme au Japon, des procédures judiciaires conduites récemment aux États-Unis à l'encontre de cadres de sociétés françaises ont montré que la dimension juridique pouvait devenir une arme de guerre économique. Que comptez-vous faire pour que notre diplomatie se donne les moyens de défendre nos entrepreneurs lorsqu'ils sont pris dans les griffes d'une « justice de l'otage », pour reprendre une expression employée par les défenseurs des droits de l'homme et par l'ONU ? La parole

vous l'avez vous-même souligné, il ne nous appartient pas de commenter la procédure judiciaire japonaise en cours. Cependant, comme il s'agit d'un Français détenu, le ministère de l'Europe et des affaires étrangères apporte naturellement son assistance à M. Carlos Ghosn au titre de la protection consulaire. Cela nous a notamment permis de nous assurer de ses conditions de détention et du respect des lois locales. Au titre de cette protection consulaire prévue par la convention de Vienne du 24 avril 1963, notre ambassade continue de lui assurer un accompagnement constant, en lien étroit

nous tenons énormément, c'est le respect de la présomption d'innocence. Le Président de la République a eu l'occasion de rappeler ces principes à l'occasion de la visite de travail en France qu'a effectuée le Premier ministre japonais Shinzo Abe Abe le 23 avril dernier. Soyez assuré, monsieur le sénateur, que nous mettons tout en oeuvre, dans le cadre de la protection consulaire, pour apporter assistance à M. Carlos Ghosn, tout en respectant évidemment la justice japonaise. La parole

Par une plus grande proximité, une meilleure réactivité, une simplification des démarches et, surtout, une personnalisation de l'accompagnement, l'école inclusive a pour objectif de sortir de l'exclusion les enfants en situation de handicap, ainsi que leurs familles.

2018-2022, qui prévoit la création d'une quarantaine d'unités sur le territoire d'ici à 2022. Madame la secrétaire d'État, je vous sais très investie dans la mise en oeuvre de ce plan doté de 344 millions d'euros. Il prévoit notamment le renforcement des unités d'enseignement pour autistes.

Le Premier ministre a mis en avant les progrès réalisés ces dernières années. En même temps, il a constaté qu'il reste énormément à faire en ce qui concerne le déploiement d'unités d'enseignement externalisées, qui permettent à ces enfants accueillis en établissement médico-social de bénéficier de l'inclusion scolaire. Madame la secrétaire d'État, comment rassurer des parents démunis, fatigués et souvent seuls ? En tant que membre de la commission des affaires sociales, je souhaiterais également savoir comment le volet médico-social du service public de l'école inclusive

a été enrichi par les travaux parlementaires. Nous devons renouer la confiance avec les familles et, surtout, mettre en avant leur expertise. Confiance, simplification et proximité sont les maîtres mots de notre démarche.

vous avez présenté mardi les mesures terribles, pour les chômeurs, de votre réforme de l'assurance chômage. Vous obéissez à l'unique obsession du Gouvernement : baisser la dépense publique ! Et pour ce faire, quoi de plus simple et de plus efficace que de sabrer dans les dépenses sociales ? Aujourd'hui l'assurance chômage, demain les retraites ma part, je veux vous parler des gens, des demandeurs d'emploi. Seuls 50 % des chômeurs inscrits à Pôle emploi bénéficient aujourd'hui d'une allocation. Parmi ceux-ci, la moitié touchent moins de 1 000 euros par mois 40 % des allocataires qui travaillent vivent dans un foyer dont les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté. Et que dire des chômeurs qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi ?

que toute personne se retrouvant au chômage puisse très rapidement être prise en charge et accompagnée vers un retour à l'emploi. Notre ambition, madame la sénatrice, est de faire en sorte que les Français puissent retrouver du travail. Cette réforme, je n'ai aucun doute à ce sujet, le permettra

Monsieur le Premier ministre, cette annonce concerne plus de 1 000 emplois directs et indirects, dans un contexte économique tendu. Elle menace également la culture de la betterave à sucre pour 2 500 planteurs et pourrait se traduire par une réduction de 10 % de que j'ai évoqués font actuellement l'objet de plusieurs scénarios de reprise mobilisant l'ensemble des agriculteurs de ces bassins. Or le groupe Südzucker ferme la porte à d'éventuels rachats. Il contourne l'esprit de la loi Florange en envisageant de laisser une poignée de salariés sur ces sites d'activité, alors qu'un plan solide de reprise a été bâti par les planteurs. Il est inadmissible que vous ne répondiez pas aux demandes d'audience que vous ont adressées dès le 29 mai les élus et les responsables de la filière. Vous renvoyez ce dossier au ministre de l'agriculture, alors que,

! Il est impératif que vous preniez les dispositions nécessaires pour favoriser le dialogue entre Südzucker et les betteraviers français. Le est inacceptable. La France ne saurait accepter une manoeuvre d'une entreprise allemande sur une partie de son industrie qui tend à casser la filière française. Que comptez-vous faire ?

Je l'ai dit au président de Südzucker il y a un mois, nous l'avons redit au numéro deux du groupe la semaine dernière : la position de cette entreprise est inacceptable pour les autorités françaises.

Ce phénomène est apparu il y a trois ans à Paris, dans le quartier de la Goutte d'Or. Depuis, il s'est progressivement étendu à la banlieue, et désormais à Bordeaux. Ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur, sans que les pouvoirs publics arrivent à l'endiguer.

Nous savons que la situation est complexe. Les mineurs étrangers sont d'abord des enfants, et ces enfants sont des victimes avant d'être des délinquants. On s'interroge encore sur l'existence de réseaux criminels qui jetteraient ces enfants dans les rues en les droguant, afin qu'ils commettent des vols pour alimenter des circuits de revente. Les associations et la justice font leur possible pour leur venir en aide. Nous ne devons pas céder au fatalisme et à la résignation. Notre responsabilité politique est d'apporter des réponses pour aider ces jeunes en errance, pour lutter contre les agressions

des résultats probants en matière de renvoi de ces mineurs dans leur pays d'origine quand un tel retour relevait de la procédure. L'action du ministre de l'intérieur s'est par ailleurs concentrée sur la lutte contre les trafics d'êtres humains, plus particulièrement sur le démantèlement des réseaux. La lutte contre les filières de passeurs, sous l'égide du parquet, est un objectif prioritaire : plus de vingt-cinq réseaux ont été démantelés en 2018. S'agissant plus particulièrement du département de la Gironde, l'arrivée de mineurs d'origine marocaine ou algérienne a en effet causé des troubles à l'ordre public. Cette arrivée est due à la modification des réseaux et des voies d'immigration en Europe.

Je vous remercie néanmoins d'avoir pris en compte la situation difficile de ces jeunes en errance. Les acteurs de terrain et les Français qui sont quotidiennement confrontés à cette misère sont relativement rassurés de voir s'amorcer un début de solution. J'espère que les élus pourront être associés à ce travail. La préfète de Gironde m'a d'ailleurs appelée à ce sujet. Il faut conclure ! Néanmoins, les acteurs de terrain et les Français qui sont quotidiennement confrontés à cette violence attendent des actes et des mesures concrètes

poignardait deux agents de l'administration pénitentiaire, au moyen d'un couteau introduit sans difficulté par sa conjointe au sein de l'enceinte carcérale. Deux jours plus tard, madame la ministre, vous nous faisiez part, dans cet hémicycle, de votre détermination à renforcer la sécurité dans les prisons par une série de mesures visant à assurer davantage d'ordre et une meilleure protection des gardiens. Trois mois plus tard, le 11 juin dernier, un détenu qualifié de « DPS », détenu particulièrement signalé, comptant à son actif cinq prises d'otages, des agressions, des viols et le meurtre d'un codétenu parvenu à prendre en otage deux surveillants pendant la distribution des repas, au moyen d'une arme artisanale fabriquée sur place. Comme le rappelait ma collègue Nathalie Goulet lors de la séance de questions d'actualité au Gouvernement du 7 mars dernier, nos prisons regorgent d'armes artisanales fabriquées par les détenus, de téléphones portables et d'armes introduites à l'occasion de visites. Force est de constater, madame la garde des sceaux, que, malgré votre détermination, le problème des armes et des portables à l'intérieur des prisons n'a toujours pas été résolu. J'entends déjà votre réponse : il est interdit aux gardiens de procéder à des fouilles systématiques et en toute circonstance des détenus et des visiteurs.

plutôt que de nous soucier de ne pas trop brusquer nos détenus, il est de notre devoir de protéger nos gardiens ? Les seules mesures que vous proposez sont d'équiper ces derniers de gilets pare-lame, de protège-cous ou de caméras embarquées. Quand vous attaquerez-vous aux causes, plutôt que d'essayer tant bien que mal de parer aux effets ?

d'État présent, M. Olivier Dussopt, m'a alors répondu en faisant référence à l'une de mes précédentes interventions, dans laquelle j'aurais parlé, selon lui, de « nocivité des contractuels », et a indiqué que le terme de « mercenaires » que j'avais employé était péjoratif et que je faisais un mauvais procès aux contractuels.

vous est donné de votre rappel au règlement, ma chère collègue. J'informe le Sénat que les candidatures pour siéger au sein de l'éventuelle commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de transformation de la fonction publique, actuellement en cours de discussion, ont été publiées. Ces candidatures seront ratifiées si la présidence n'a pas reçu d'opposition dans le délai d'une heure prévue par notre règlement.

le rapport d'information intitulé « Donner un nouveau souffle à la politique du handicap dans la fonction publique », que mon collègue Didier Marie et moi-même avons rédigé. Le texte de la commission reprend plusieurs propositions de ce rapport afin de mieux intégrer les agents en situation de handicap et de pérenniser le financement de cette politique.

pouvant recourir au recrutement par contrat. Actuellement, le recours au contrat pour certains emplois est possible pour les intercommunalités dont la population moyenne par commune est inférieure à 1 000 habitants. Cette rédaction permet à une intercommunalité de 50 000 habitants comptant cinquante et une communes de bénéficier de cette faculté. Or le recours au contrat a vocation à concerner en priorité les petites communes ou les petits groupements, qui ont des difficultés à attirer des agents. Un groupement de plus de 50 000 habitants n'entre à l'évidence pas dans ce cadre. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale, des amendements similaires de plusieurs groupes, dont un du groupe socialiste, a limité le recours au contrat aux intercommunalités comptant jusqu'à 15 000 habitants. Cet amendement vise à conserver cette mesure. Pour le reste, il tend à supprimer les principales dispositions de l'article qui élargissent les possibilités de recourir au contrat dans la fonction publique territoriale. Nous avons dit hier soir tout le bien que nous pensions de cette extension excessive du champ du recours au contrat ...

Si une telle modification est louable, le seuil retenu ne paraît pas opportun. En effet, de nombreuses communes dont la population est juste supérieure à ce seuil se verraient exclues du dispositif, alors même qu'elles en ont un besoin extrêmement important. Le mouvement de regroupement de communes observé ces dernières années amplifie cette situation, sans être pris en compte par le projet de loi. Avec un plafond fixé à 2 000 habitants, un important effet de seuil se ferait sans doute ressentir. égard au besoin exprimé par de nombreux maires d'avoir recours au contrat pour pourvoir des postes vacants, il nous semble intéressant de relever le seuil. C'est pourquoi le présent amendement tend à autoriser le recrutement pour tous les emplois de contractuel dans les communes de moins de 5 000 habitants.

que le recours au contrat soit possible dans les intercommunalités de moins de 50 000 habitants. Un grand nombre de députés ont proposé de limiter la taille des intercommunalités concernées à 15 000 habitants. Un amendement en ce sens a été adopté avec un avis favorable du Gouvernement.

Cela revient à augmenter très fortement le nombre de communes concernées par la possibilité de recrutement indifférencié par contrat, indépendamment des autres possibilités ouvertes par le projet de loi,

les territoires ruraux. Ce faisant, sous prétexte d'élargir le vivier de recrutement, vous introduisez une inégalité territoriale flagrante. Enfin, vous permettez

permet pourtant de garantir aux collectivités employeurs, sur l'ensemble du territoire, quelle que soit leur taille, un haut niveau de compétence, certifié par des concours aux référentiels nationaux : c'est l'égalité républicaine.

122 rectifié vise à supprimer l'essentiel des dispositions de l'article 10, qui apporte pourtant des assouplissements bienvenus aux règles de recrutement d'agents contractuels par les employeurs publics territoriaux. La commission a donc émis un avis défavorable.

La dérogation dont bénéficient les petites communes se justifie par le fait qu'il s'agit souvent d'emplois à temps partiel, voire très partiel, ne nécessitant pas une formation initiale particulière.

le concours ouvre le droit à l'affectation et, dans le cas d'un nombre insuffisant de postes, une liste d'attente est établie ; une fois cette dernière épuisée, si de nouveaux besoins apparaissent, les administrations peuvent alors recourir au contrat. Cela semble plutôt relever du bon sens, puisqu'il s'agit de lancer la carrière d'une personne ayant prouvé, par la réussite à un concours, sa capacité à occuper un emploi public.

en cas de postes insuffisants, une liste complémentaire est créée et elle doit être épuisée avant tout recrutement hors statut. Pour la fonction publique territoriale, le système est effectivement un peu différent, puisque l'inscription sur une liste d'aptitude vaut non pas recrutement, mais seulement reconnaissance du droit à l'embauche. Toutefois, l'essentiel est bien là la liste d'aptitude est un gage, tant pour les agents que pour les collectivités, que les inscrits ont toutes les compétences pour pourvoir à des postes vacants. Par ailleurs, ayant une valeur nationale, cette liste permet à l'ensemble des collectivités territoriales de faire des propositions d'embauche.

qui mériterait une publicité plus importante. Cet amendement vise donc à rappeler ce qui fait à nos yeux la base même de l'accès à la fonction publique : la réussite à un concours. Il tend ainsi à encadrer le recours aux contractuels en donnant priorité aux fonctionnaires. Cela offre une sécurité aux lauréats des concours, mais c'est aussi l'assurance, pour les administrations employeuses,

l'avis de la commission ? Les employeurs publics territoriaux sont aujourd'hui habilités à recruter des agents contractuels pour une durée d'un an renouvelable, afin de faire face à une vacance temporaire d'emploi, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Nos collègues proposent de préciser que cette faculté ne pourra être exercée que lorsque la liste d'aptitude correspondante est épuisée. J'y vois deux écueils. premier lieu, il existe non pas une seule liste d'aptitude, mais autant de listes d'aptitude que de concours. Un employeur public territorial peut très bien recruter un agent qui a été admis à un concours organisé à l'autre bout de la France, par un centre de gestion dont il ne relève pas.

de l'amendement aboutirait à lier les mains de l'autorité territoriale, qui, le cas échéant, serait forcée de recruter le dernier candidat inscrit sur une liste d'aptitude, quand bien même celui-ci ne lui semblerait pas adapté à l'emploi à pourvoir.

Je tiens à préserver le principe selon lequel la nomination dans les emplois de la fonction publique territoriale est de la compétence exclusive des autorités territoriales. La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Cet amendement vise à préciser le cadre applicable à une situation très spécifique, que rencontrent à vrai dire de nombreux employeurs locaux : il s'agit du cas d'agents contractuels recrutés dans un certain cadre d'emploi où est susceptible d'intervenir un agent titulaire. Ce dernier peut souhaiter passer d'un temps non complet à un temps plein. Le Conseil d'État a jugé le 19 décembre 2018 une affaire dans laquelle une collectivité avait refusé à un agent titulaire la possibilité de bénéficier d'un temps complet, tout en ayant recruté un agent contractuel pour intervenir sur les mêmes fonctions. Le Conseil d'État a estimé que la collectivité aurait dû accepter la demande de passage à temps complet de l'agent titulaire. Dit autrement, le recrutement d'un agent contractuel ne peut, dans ce cas, intervenir qu'à titre complémentaire. Cet amendement tend donc à apporter une garantie supplémentaire aux fonctionnaires. Mais cette disposition est aussi conditionnée aux exigences d'organisation du service et au besoin des services, c'est-à-dire qu'elle ne sera pas applicable à la situation où le fonctionnaire en question n'est pas disponible sur les horaires du service complémentaire. Vous le voyez, mes chers collègues, cet amendement vise à apporter une certaine sécurité juridique aux collectivités locales dans ce type de situation, raison pour laquelle je vous demande de le voter. Quel est l'avis de la commission ? ? Cet amendement tend en effet à s'inspirer d'une décision du Conseil d'État du 19 décembre 2018, dans laquelle la haute juridiction a enjoint à la communauté d'agglomération de Toulon de nommer à temps complet un professeur d'enseignement artistique qui en faisait la demande, demande que la communauté d'agglomération avait rejetée, alors même qu'elle avait recruté un agent contractuel à temps partiel pour enseigner dans la même discipline. En l'occurrence, les besoins du service ne justifiaient pas d'avoir recours à un agent contractuel. L'amendement a pour objet de légaliser cette jurisprudence, ce qui ne soulève pas d'objection de principe, même si cela ne ferait pas forcément évoluer le droit positif.

notamment des aides-soignants et des infirmiers. Cette situation est due en partie au fait que l'exercice de cette profession nécessite d'obtenir un diplôme d'État, mais également de réussir à un concours de la fonction publique territoriale. Ce mode de recrutement ne s'applique pas dans les établissements de statut différent, qu'ils soient privés, associatifs la fonction publique hospitalière. Ces derniers recrutent directement leur personnel à partir des diplômes professionnels d'État. Alors qu'ils manquent cruellement d'aides-soignants et d'infirmiers, le recours obligatoire à un concours spécifique est particulièrement pénalisant et discriminatoire pour les établissements relevant de la fonction publique territoriale. Cela les conduit fréquemment à faire appel, dans l'urgence, à l'intérim pour assurer des soins aux personnes âgées. Cette situation suscite des coûts supplémentaires pour les résidents, souvent de condition modeste, mais aussi pour les budgets publics. Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi du 26 loi du 26 janvier 1984 portant diverses dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, afin de dispenser de concours les aides-soignants et infirmiers qui souhaitent travailler dans un Ehpad public territorial. Cette dispense permettrait d'aligner le recrutement des Ehpad publics territoriaux sur le recrutement des autres établissements. C'est une nécessité urgente pour améliorer les conditions de vie de nos aînés, mais aussi pour faciliter le recrutement de ces

parce que, dans la fonction publique territoriale, les fonctionnaires des filières sociales, médico-sociales et médico-techniques peuvent être recrutés au moyen d'un concours sur titre. Il est donc possible de recruter des infirmiers, par exemple, par le biais du concours sur titre,

Je ne prendrai qu'un exemple : comment la Ville de Lyon a-t-elle pu mettre plus de trois ans pour procéder au recrutement d'un directeur général des services, alors même que des candidats lui étaient proposés par le maire d'arrondissement concerné ?

Cette question est d'autant plus légitime que la mutation que les différents gouvernements ont imposée à la fonction publique, avec un retour des liens hiérarchiques forts entre pouvoir politique et administration n'invite vraiment pas les agents à aller devant les tribunaux, de peur de peur de voir leur carrière brisée. Deuxièmement, j'ai bien du mal à me satisfaire d'une procédure contentieuse de plus de sept ans, qui a porté préjudice au plaignant. Il me semble qu'il faut aussi s'interroger sur l'intérêt qu'éprouvent les collectivités à recourir à l'emploi intérimaire. Clairement, ce dernier n'est pas économiquement favorable,

La deuxième, qui est problématique, consiste à recruter sur un temps très court des intérimaires pour assurer le service minimum en cas de grève et donc remplacer les grévistes- il est tout de même étonnant, alors que le Gouvernement manifeste sa volonté de rapprocher le secteur public du secteur privé, qu'il maintienne légal dans la fonction publique ce qui ne l'est pas dans le privé, en application de l'article L. 1251-10 du code du travail. La troisième, tout aussi problématique, est que les collectivités peuvent ainsi abandonner leurs obligations d'employeur en les déléguant totalement à des entreprises régulièrement épinglées pour leur manque de respect pour la législation du travail, ce qui pose d'ailleurs la question du règlement des conflits en contentieux, puisque si la juridiction administrative a jusqu'ici pris en charge ces dossiers, ce n'est pas forcément naturel. Quel est l'avis de la commission ?

Je rappelle que le recours à l'intérim est doublement encadré. Par le droit, tout d'abord, la loi définissant les situations justifiant de faire appel à un intérimaire- besoin occasionnel, remplacement imprévu, etc. Les employeurs territoriaux doivent d'ailleurs faire appel aux services de remplacement des centres de gestion, avant de pouvoir recourir à l'intérim.

D'après les informations recueillies lors de l'examen de la loi Déontologie, le recours à l'intérim reste peu fréquent : seul 1,5 % des collectivités territoriales font appel à des intérimaires. Dans la fonction publique d'État, l'intérim représente moins de 150 équivalents L'intérim est plus important dans la fonction publique hospitalière, pour assurer la continuité du service. Conservons cette souplesse

Hélas, devant la pénurie de médecins hospitaliers, les établissements n'ont souvent d'autre choix que de recourir à l'intérim. Nous le vivons tous dans nos territoires. En moyenne, une journée de travail pour un médecin intérimaire lui rapporte entre 600 et 800 euros nets, soit un coût de 1 370 euros TTC pour l'hôpital, c'est-à-dire le triple du coût normal d'une journée de travail par rapport à un médecin titulaire. Ce recours massif à des médecins remplaçants- que l'on peut tout de même qualifier d'« hors de prix » -concerne toutes les spécialités médicales,

Un amendement a été adopté au Sénat lors de l'examen de la loi Santé pour un meilleur encadrement des écarts de rémunération entre les personnels titulaires et contractuels, afin de lutter contre l'intérim médical, en attendant les résultats de la concertation au ministère de la santé à restaurer l'attractivité des postes de médecin hospitalier. Toutefois, le refus de la ministre d'évoquer la question de la hausse des salaires risque, à notre avis- nous nous trompons peut-être -, d'entraîner la négociation dans une impasse. En attendant, l'intérim reste un fléau dans la fonction publique hospitalière, qui a dû réaliser-

cette situation est préjudiciable au bon fonctionnement des services ; en tout cas, elle est source d'iniquité entre les agents, car il n'y a pas de raison que, pour des fonctions similaires,

est le sens de cet amendement. en imposant au pouvoir réglementaire de définir un statut d'emploi commun pour tout « ensemble de situations de travail caractérisé par des activités identiques ou fortement semblables ». Or il tend à modifier la loi du 26 janvier 1984, qui concerne non

cela rejoint votre souhait -à la fois une meilleure coordination interministérielle entre les différents corps, pour garantir une forme d'égalité, et le maintien de conditions d'emploi non statutaires, plutôt en matière indemnitaire ou d'avantages particuliers liés au rattachement ministériel. Il existe un certain nombre d'exemples assez frappants. Dans des départements de petite ou moyenne taille, selon le point de vue, qui comptent entre 300 000 et 400 000 habitants, les directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations, peuvent accueillir entre 80 et 100 agents qui, ce n'est pas rare, peuvent dépendre de 14 ou de 15 budgets opérationnels de programme, ou BOP, donc d'autant de conditions différentes pour tel ou tel aspect de leur carrière ou de leur rémunération. Ce matin se tenait un comité interministériel de la transformation publique qui a été l'occasion pour le Premier ministre d'annoncer le rapprochement de certains services déconcentrés, ainsi que la volonté de mutualiser les fonctions support, notamment au niveau des secrétariats généraux. Pour ce qui me concerne, j'ai appelé appelé mes collègues à saisir et les secrétaires généraux des ministères et les responsables des services déconcentrés, pour que, chaque fois que c'est possible, nous puissions rapprocher ou fusionner ces fameux BOP- pardonnez-moi ce sigle -et faire en sorte que, dans les services déconcentrés et les fameuses directions interministérielles,

Nous avons tenu en effet à compléter la liste des causes d'indisponibilité justifiant d'avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible, en y incluant l'ensemble des congés qui peuvent être accordés aux fonctionnaires territoriaux. En effet, cette liste est aujourd'hui à la fois incomplète et obsolète, pour la seule raison que l'on a oublié de l'actualiser, lorsqu'on a créé de nouveaux congés ou modifié les congés existants. Nous y avons aussi inclus certains cas de détachement et de disponibilité, en ciblant précisément les cas dans lesquels le fonctionnaire détaché ou placé en disponibilité ne peut être remplacé, et où il doit, à l'issue de cette position, être réintégré dans son emploi. Cela justifie pleinement à nos yeux qu'il soit fait appel un agent contractuel pour le remplacer temporairement. La commission émet donc un avis défavorable.

pour notre part que la commission a élargi inconsidérément les possibilités de recrutement de contractuels pour suppléer

au service civique, nous paraît excessif. Même si nous considérons qu'il est légitime que le Sénat, qui représente les collectivités territoriales, réponde aux besoins exprimés par les employeurs territoriaux, nous ne souhaitons pas, dans l'esprit d'ailleurs de ce que nous avons défendu jusqu'à présent, libéraliser à outrance les recrutements sur contrat et donc ignorer le sort des fonctionnaires territoriaux, c'est-à-dire celles et ceux qui ont fait le choix de passer des concours pour s'engager auprès de ces mêmes collectivités. Il doit être possible de trouver des solutions alternatives au contrat pour les remplacements concernés. ? Quel est l'avis de la commission ?

n° 138 rectifié . Cet amendement a pour objet d'ajouter le congé pour invalidité temporaire imputable au service à la liste des motifs qui justifient, dans la fonction publique territoriale, d'avoir recours à un agent contractuel pour remplacer un agent momentanément indisponible. S'agissant

Étant donné l'état d'épuisement de l'ensemble du personnel de nos hôpitaux, cette décision nous paraît particulièrement inappropriée. Comme dans le secteur privé, où désormais CDD sur dix sont d'une durée inférieure à un mois, l'effet d'aubaine anticipé est fortement contestable. Il semble plutôt se situer du côté des employeurs, lesquels sont en position de force face à des employés captifs et bon marché. Après l'annonce pour les recours abusifs aux contrats courts, et à l'approche de la réforme de l'assurance chômage, il serait incohérent de prévoir des facilités pour les employeurs publics hospitaliers. C'est la raison pour laquelle nous défendons le rétablissement

L'Assemblée nationale a adopté un dispositif permettant de créer une prime de précarité dans les trois versants de la fonction publique pour les contrats d'un an ou moins, à l'exception des contrats saisonniers.

pour assurer la continuité des soins nous oblige à limiter l'application de la prime de précarité, afin de ne pas aggraver l'état financier des établissements. » Le Gouvernement étant à l'origine de cette disposition, il va sans dire qu'il va financer les 400 millions d'euros et garantir le financement de cette prime de précarité aux hôpitaux. M. le secrétaire d'État pourra nous le confirmer.

À défaut, cette prime semblerait absolument inéquitable et créerait une inégalité entre les différentes fonctions publiques, ce qui est contraire à l'esprit du statut. Mes chers collègues, nous demandons, en conséquence, le rétablissement du texte

la commission a entendu prendre en compte la situation particulière des hôpitaux, en excluant du champ de cette prime les personnels recrutés pour remplacer un agent indisponible, faire face à une vacance d'emploi ou à un accroissement temporaire d'activité.

particuliers et que les hôpitaux français sont dans une situation financière déplorable. Dans ces conditions, que faut-il faire ? Au nom d'une idée généreuse, étendre la nouvelle prime de précarité à l'ensemble des agents contractuels hospitaliers ?

le périmètre de la mesure, un souci d'équité envers les autres fonctions publiques et le secteur privé qui me convient. Plusieurs de nos collègues ont dit qu'il fallait faire pour la fonction publique hospitalière ce que l'on s'apprête à faire pour le secteur privé dans le cadre de la réforme de l'assurance chômage et ce que l'on a déjà décidé de faire pour la fonction publique de l'État et la fonction publique territoriale. Si nous devons aller dans cette direction, malgré cette source d'insatisfaction qui demeure, alors il faut faire ce que vous nous proposez.

visait à supprimer l'obligation faite aux employeurs publics territoriaux de nommer en tant que fonctionnaires stagiaires leurs agents contractuels admis à un concours de la fonction publique territoriale et inscrits sur une liste d'aptitude.

placer demain les agents publics contractuels dans une démarche de construction de compétences, par l'accès au concours, si la réussite à ce dernier n'aboutit pas à une titularisation ?

de renforcer une équipe ou de s'assurer, par le biais du contrat, que la personne qu'il recrute dispose des compétences requises pour assurer le service. Cet agent, en cours de mission, passe un concours et le réussit.

des agents contractuels publics en CDD à obtenir leur « CDIsation », ainsi que les nombreux cas de recours abusifs à des CDD, qui ne donnent lieu ni à des requalifications, quand ces cas sont portés devant le Conseil d'État, ni à des sanctions à l'encontre des employeurs se plaçant dans l'illégalité. À la lumière de ce constat, nous considérons donc que des passerelles devraient être aménagées du statut contractuel vers celui de fonctionnaire, afin de mieux reconnaître et de mieux récompenser l'engagement continu d'un agent pour le service public. Dans cet esprit, cet amendement vise à rétablir

en matière sociale et économique avait pour objectif de faciliter les demandes de mutation émises par les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux, dans l'une des collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution. Ces intérêts matériels et moraux devaient donc constituer une priorité à prendre en compte par l'administration lors d'une demande de mutation, quel que soit le corps d'origine du fonctionnaire. Force est de constater, et vous le savez bien monsieur le secrétaire d'État, qu'il s'agit d'un échec : cette loi n'est tout simplement pas appliquée au sein de la fonction publique, notamment de la police nationale, dans laquelle un seul poste sur quatre est réservé à un agent

dure réalité quotidienne est la suivante pour nos fonctionnaires ultramarins : demande après demande, année après année, leur administration refuse qu'ils rentrent chez eux dans le cadre de leur mutation. On leur oppose une nécessaire modification de l'outil informatique permettant le calcul des points

Il s'agit ni plus ni moins d'un véritable scandale à l'égard de nos fonctionnaires ultramarins, qu'ils soient de Martinique, de La Réunion, de la Guadeloupe, etc., d'autant que la jurisprudence et les administrations ont réduit, au fil des années, le champ d'application de la notion du CIMM. Nos concitoyens fonctionnaires massivement affectés dans l'Hexagone se voient donc systématiquement refuser leurs mutations et leurs congés bonifiés. Cela doit cesser ! C'est pourquoi je voterai les amendements déposés par mes collègues sur ces sujets. La parole

Le Gouvernement développe un argumentaire selon lequel cela permettra d'accélérer les nouvelles affectations. On peut toutefois se demander si les comités sociaux nouvellement créés auront un réel pouvoir sur la définition des lignes directrices de gestion en matière de mobilité.

permettaient de mettre de l'huile dans les rouages de la machine administrative, en venant éclairer le choix de l'employeur public par une bonne connaissance des dossiers, voire par la correction de barèmes mal renseignés.

J'attire votre attention, également, sur la problématique tout aussi préoccupante des enseignants qui passent des concours au niveau master et qui sont contraints de venir systématiquement dans l'Hexagone, sans possibilité de rentrer, la plupart du temps, dans leurs différents territoires

de loi. Ici, vous renforcez non seulement l'arbitraire de l'administration sur les décisions individuelles relatives aux mutations des agents, mais aussi la dépendance des agents envers leur hiérarchie,

favoriser les pressions ou les comportements clientélistes. Alors même que vous ne cessez, depuis le début de l'examen de ce projet de loi, de répéter à qui veut l'entendre que vous promouvez

En quoi le fait de supprimer l'avis des commissions administratives paritaires renforce-t-il le dialogue entre l'administration et les représentants des agents ? En quoi l'avis de ces commissions est-il un frein aux procédures de mutation des agents ? Enfin, qui demande de

Jasmin et M. Antiste. Pour le reste, nous considérons que supprimer l'examen des situations individuelles par la CAP permettra effectivement de gagner du temps et que la définition des règles d'accès à la mobilité dans le cadre des lignes directrices de gestion, ainsi que le droit de recours qui a déjà été voté, garantira l'équité. Il faut avoir en tête que, en matière de fonction publique d'État dans les services déconcentrés, lorsqu'un chef de service doit faire face à un départ inopiné, s'il souhaite recruter

toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service », quelques priorités, lesquelles, à la lecture de l'article, ne seront cependant pas opposables. Il s'agit d'une remise en cause majeure du dialogue social, de la capacité des délégués à défendre les agents

nous considérons qu'exclure des compétences des CAP la question des mutations est un choix funeste et une mauvaise manière envers les personnels.

est à M. Maurice Antiste. La qualité du service rendu dépend beaucoup du bien-être des agents dans leur travail ; honorer leur demande d'affectation ne peut qu'y contribuer.

Jérôme Durain. Cet amendement tend à supprimer une mention qui restreint la priorité de mutation pour les couples pacsés séparés pour des raisons professionnelles. En effet, le fonctionnaire pacsé ne peut bénéficier d'une priorité de mutation que s'il produit la preuve que son couple se soumet à l'obligation d'imposition commune prévue à l'article 6 du code général des impôts. Sont donc exclus de cette priorité de mutation, les pacsés qui optent pour le régime dérogatoire de la séparation de biens. Or ce régime est généralement admis pour les couples disposant de deux domiciles séparés, notamment pour des raisons professionnelles. Les exclure des demandes de priorité permettant la réunion du couple nous paraît dès lors constituer un contresens. Les deux amendements suivants sont identiques. L'amendement n° 241 rectifié

Pourtant, près de deux ans après l'entrée en vigueur de cet article, précisé par la circulaire du 1 mars 2017, les fonctionnaires et leurs représentants signalent de nombreux dysfonctionnements quant à son application.

Nous souhaitons également rappeler que les demandes de mutation et les questions de mobilité sont exclues des prérogatives des commissions administratives paritaires et reviennent donc aux services des ressources humaines des administrations,

Deux ans après l'entrée en vigueur de ces dispositions, précisées par une circulaire du 1 mars 2017, les syndicats de fonctionnaires ultramarins ne cessent de signaler de nombreux dysfonctionnements quant à leur application.

Depuis la loi de programmation relative à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique, la loi ÉROM, celle-ci a une valeur légale et concerne tous les fonctionnaires, quels que soient leurs corps,

Le retour des fonctionnaires originaires des outre-mer dans leur territoire est un enjeu majeur. En effet, de nombreux fonctionnaires ultramarins présents dans l'hexagone attendent souvent des années un retour qui ne vient parfois jamais. Ils vivent des situations de détresse extrême, en étant parfois séparés par des milliers de kilomètres de leur famille ou de leurs parents dépendants. Par ailleurs, la Martinique et la Guadeloupe connaissent un effondrement démographique sans précédent et sans équivalent ailleurs en France. La Martinique, par exemple, perd dix habitants par jour en moyenne. Depuis dix ans, sa population a baissé de 8 %. La collectivité comptait près de 400 000 habitants en 2010 et, si la tendance se poursuit, elle n'en comptera plus que 280 000 en 2050, selon une estimation de l'Insee.

des instituts régionaux d'administration, les IRA, le bénéfice des dispositions de la loi ÉROM relatives à la prise en compte des centres d'intérêts matériels et moraux, afin de leur permettre une première affectation dans leur territoire d'origine. Il s'agit de faire respecter, dès l'entrée en fonction des nouveaux agents, ce droit inhérent aux fonctionnaires venant d'outre-mer, qui attendent bien souvent de trop longues années avant de pouvoir être mutés dans leur territoire d'origine. Il nous semble regrettable que de nombreux jeunes fonctionnaires, dont le coeur de métier sera en rapport avec les spécificités territoriales de leur affectation, ne puissent pas faire profiter l'administration qu'ils serviront de leur expérience et de leur expertise. Les instituts régionaux d'administration forment des fonctionnaires qui joueront un rôle d'encadrement et de direction important de futurs cadres de la fonction publique, qui devront se montrer moteurs dans les administrations. Un attachement préalable à un territoire, à ses habitants et à ses pratiques nous paraît d'excellent augure pour la conduite de ces missions. De même, nous pensons que l'éloignement du territoire d'origine et toutes les difficultés qui peuvent en résulter ne sont pas de nature à favoriser les débuts dans leurs fonctions de ces agents, ni leur futur parcours professionnel.

En effet, s'agissant d'égalité réelle, il est peu concevable que des disparités d'application induisent une inégalité de traitement des agents au sein de certains ministères. Il devient urgent que toutes les administrations de l'État puissent se référer aux mêmes critères, pour prévenir toute rupture d'égalité d'un ministère à l'autre. Il s'agit, une fois de plus, de faire de la transparence et de l'équité des valeurs sur lesquelles tous les agents publics peuvent compter, des valeurs propres à lever l'ensemble des doutes et des craintes des fonctionnaires et de leurs représentants.

signataire, vise à obliger les employeurs publics à procéder à un classement préalable des demandes de mutation à l'aide d'un barème rendu public et commun à l'ensemble de la fonction publique

une nouvelle rigidité, cette mesure mettrait un terme aux rigidités organisées par certains employeurs publics.

devant être pris en considération pour identifier l'existence d'un tel centre. Il est indispensable que les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux soient précis et d'application générale à toutes les administrations concernées. Selon les chiffres fournis par le ministère de la fonction publique lors de l'examen du présent projet de loi à l'Assemblée nationale, quelque 27 % des demandes de mutation outre-mer ne seraient pas satisfaites, et les agents ayant déposé des demandes avant la promulgation de la loi ÉROM sont tenus de déposer de nouveau un dossier faisant mention du CIMM. Cet amendement vise à garantir l'égalité de traitement et la sécurité juridique dans le traitement des demandes de mutation présentées en raison de l'existence d'un centre des intérêts matériels et moraux outre-mer. Une telle précision semble nécessaire, puisque, à la suite de la décision du ministère de l'intérieur de reporter de quelques mois la prise en compte de l'existence des CIMM pour les mutations de policiers, le Conseil d'État a dû rappeler, par un arrêt du 18 mars dernier, que la priorité légale d'affectation liée à l'existence d'un centre des intérêts matériels et moraux dans un territoire ultramarin était d'application immédiate et générale.

outre-mer. Il est indispensable que les critères de détermination des centres des intérêts matériels et moraux soient précis et d'application générale à toutes les administrations concernées par le présent projet

Comme le souligne la circulaire du 1 mars 2017, la création des centres des intérêts matériels et moraux est une étape majeure dans la prise en compte de la situation spécifique des fonctionnaires ultramarins de l'État. dispositions des nombreux amendements déposés montrent qu'il existe un réel problème de clarté et d'homogénéité dans la définition et l'application de cette notion. Pour l'heure, les seuls critères ont émergé de la jurisprudence administrative et ont été rassemblés dans une circulaire.

est favorable sur les amendements identiques n 241 rectifié de Mme Assassi et 424 rectifié de M. Lurel. Comme nous le verrons après l'article 11, nous sommes exceptionnellement favorables, monsieur

L'amendement n° 88 rectifié, de Mme Conconne, vise à donner une priorité systématique aux mutations de fonctionnaires d'État dont le centre des intérêts matériels et moraux est outre-mer.

part, à la sortie des IRA, les fonctionnaires stagiaires sont non pas mutés, mais affectés. D'autre part, cette affectation est prononcée en fonction des choix des élèves et de leur classement de sortie. Il semble donc difficile d'y intégrer les priorités prévues en matière de mutation.

supprimer la mention selon laquelle les couples pacsés doivent se soumettre à une obligation d'imposition commune pour bénéficier d'une priorité dans les choix de mutation. Nous sommes bien évidemment en faveur d'une plus grande égalité dans le rapprochement familial, mais nous craignons que cette modification technique n'entraîne un retour au PACS à cette seule fin et en détourne l'objet. Nous demandons l'avis du Gouvernement, qui nous dira si un tel risque est possible du fait de cette seule modification. modification. Les amendements n 136 rectifié de M. Lurel et 243 de Mme Assassi, quasiment identiques, tendent à ce que le barème sur lequel l'administration doit se fonder pour prononcer les mutations soit commun à toute la fonction publique d'État. devant la diversité des profils, des emplois et des besoins de la fonction publique à l'échelle de tout le territoire, il semble impossible de créer un tel barème unique. On ne peut pas affecter avec les mêmes critères un agent de catégorie C et un jeune inspecteur des finances, par exemple.

Avec son amendement n° 132 rectifié , M. Durain propose de supprimer la nécessité de fournir une preuve de l'imposition commune pour les couples pacsés demandant à bénéficier d'une priorité de mutation.

n'est ouverte que pour les revenus acquis au titre de la première année du PACS. Inversement, en dehors de la première année du PACS, l'imposition séparée est possible pour les couples séparés de biens et ne vivant pas sous le même toit, en cas d'instance de séparation de corps ou de divorce, lorsque le couple a été autorisé à avoir des résidences séparées, et en cas d'abandon du domicile conjugal par l'un ou l'autre des époux ou des pacsés, lorsque chacun dispose de revenus professionnels ou patrimoniaux distincts, en application du 4° de l'article 6 du code général des impôts.

permet, d'une certaine manière, de passer devant d'autres agents qui souhaitent la même mutation, nous trouvons opportun de maintenir un véritable contrôle de la réalité du couple, donc de la nécessité du rapprochement.

Positif, parce que, au risque de surprendre les parlementaires ultramarins, quelque 75 % des demandes de mutation déposées au titre de l'année 2018 par des fonctionnaires bénéficiant d'un CIMM ont été suivies d'une mutation correspondant au voeu

cette priorité légale d'affectation s'entend uniquement s'il est ouvert un poste correspondant aux qualifications, aux compétences et au grade de l'agent qui y prétend. Qu'aucun poste ne soit ouvert est effectivement un frein à l'application du CIMM. La nomination d'un élève

du Gouvernement, de permettre l'organisation de concours nationaux à affectation locale, ce qui permettra notamment à certains de nos concitoyens originaires d'outre-mer de se présenter à des concours nationaux en ayant la certitude d'être affectés

serait certainement moins protecteur, en tout cas moins englobant, que le recours jurisprudentiel à un faisceau d'indices permettant d'avoir une appréciation plus souple

d'expérience, je sais que c'est un peu à la bonne volonté du fonctionnaire qui décide- c'est triste à dire, mais c'est ainsi. Nous sommes là pour faire la loi, et je ne comprends pas pourquoi, puisque l'occasion nous en est donnée, nous ne réglerions pas les problèmes de flou.

de créer dans certains territoires d'outre-mer une direction unique des ressources humaines mutualisant les compétences en matière de ressources humaines pour plusieurs ministères. Les territoires concernés sont Wallis-et-Futuna, La faculté de mobilité entre les services regroupés au sein de la direction unique étant encadrée par la définition d'une règle de priorité de mutation au bénéfice des agents de l'État déjà affectés dans la collectivité, les conditions et proportions de postes ouverts

qui sont déjà affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps, de corps. La priorité légale interviendrait désormais sans distinction selon que la mutation s'opère, ou non, selon un tableau périodique de mutation. La mention de cette procédure est en réalité sans incidence sur la portée de la priorité légale.

de la loi du 28 février 2017 s'agissant de la mise en place d'une direction unique des ressources humaines pour l'État dans les territoires de Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Wallis-et-Futuna, en tenant compte des évolutions apportées en matière de gestion des ressources humaines par le présent projet de loi. Ces dispositions reconnaissent aux agents publics placés sous l'autorité du représentant de l'État qui sont déjà affectés à Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou Wallis-et-Futuna, ainsi qu'aux agents déjà en fonction sur le territoire concerné qui bénéficient d'un avancement de grade ou d'une promotion de corps, une priorité de mutation pour pourvoir les postes vacants dans les services de l'État sur ces territoires. Cette priorité légale interviendra désormais sans distinction selon que les mutations s'opèrent ou non selon un tableau périodique de mutation.

Mme Éliane Assassi. Transparence, adaptabilité et effectivité du droit sont des notions soeurs. C'est particulièrement vrai pour les matières qui nous intéressent ici, à savoir les mutations de fonctionnaires. Les agents publics issus des territoires ultramarins sont régulièrement confrontés à des situations d'une difficulté particulière, tendant à leur éloignement de leurs régions et départements À cette fin, sur la base de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, l'article 85 de la loi du 28 février 2017 a instauré une priorité dans les mouvements de mutation pour les fonctionnaires qui justifient du centre de leurs intérêts matériels et moraux dans un territoire d'origine.

de nombreux dysfonctionnements ont été signalés par les syndicats d'agents publics dans l'application du mécanisme institué par la loi du 28 février 2017. Il paraît donc pertinent que le Gouvernement produise un rapport

s'inscrirait dans la tendance actuelle visant une meilleure adaptabilité du droit public aux usagers, mais également aux agents. Elle permettrait enfin à la représentation nationale, mais également au Gouvernement, de définir les pistes nécessaires à l'évolution du cadre juridique actuel.

Il est donc important que les chefs d'établissement aient leur mot à dire sur les personnels qui sont affectés dans leur établissement, afin de garantir la meilleure adéquation possible entre le profil du candidat et le projet de l'établissement ou le poste proposé. Outre les postes à profil, il est donc prévu que le chef d'établissement soit systématiquement associé aux décisions d'affectation des enseignants et des personnels d'éducation qui sont nommés dans son établissement, comme c'est d'ailleurs le cas pour les professeurs des établissements privés sous contrat. L'amendement privés sous contrat. L'amendement n° 200 rectifié est le fruit de discussions que nous avons déjà eues. Un certain nombre d'enseignants chevronnés et dotés d'une solide expérience se déclarent prêts à exercer dans un établissement plus difficile.

objet d'instituer un mode d'affectation dérogatoire au mouvement au barème, fondé sur une logique d'engagement réciproque : un enseignant expérimenté accepte d'exercer pendant une durée déterminée des fonctions dans un établissement appartenant à une liste fixée par le recteur, et l'institution s'engage à ce qu'il retrouve son poste ou un poste comparable dans son établissement d'origine ou, à défaut, dans un établissement comparable de la même ville ou du même secteur.

que nous sommes parfois confrontés à un dans l'affectation des agents du ministère de l'éducation nationale. En effet, le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré précise que ces derniers peuvent être affectés « exceptionnellement dans les classes de collège ».

parce que leur plus-value disciplinaire les destine naturellement au lycée, aux classes préparatoires aux grandes écoles ou à l'enseignement supérieur, comme l'a rappelé plusieurs fois la Cour des comptes. Nous demandons donc, au travers de cet amendement, un rapport au Gouvernement

l'affectation d'un enseignant pourrait procéder d'un engagement réciproque conclu avec l'autorité de l'État responsable en matière d'éducation pour une durée déterminée, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Or les modifications apportées par l'article 11 du projet de loi aux règles applicables en matière de mutation dans la fonction publique d'État ouvrent déjà cette possibilité, en prévoyant que l'autorité compétente pourra définir, dans des conditions prévues

aujourd'hui. Sur le fond, nous nous opposons à cette mesure, qui nous paraît extrêmement dangereuse. La politique d'affectation doit rester nationale. Le système est déjà extrêmement perverti par la combinaison de l'établissement de la carte scolaire et du choix des options et spécialités. Il permet aux familles de contourner la carte, ce qui concourt à la création d'établissements élitistes et d'établissements ghettos ! En donnant un droit de regard sur les nominations aux chefs d'établissements, ce phénomène se trouvera renforcé : il y aura les « bons » et les « mauvais » personnels, comme il y a déjà les « bons » et les « mauvais » établissements. On imagine assez aisément les pressions qui seront exercées sur les chefs d'établissements. Les questions de personnes vont entrer en ligne de compte dans la politique d'affectation ... Je vous laisse imaginer l'atmosphère

éprouvent d'immenses difficultés à revenir, lorsqu'ils en font la demande, au sein de leur territoire d'origine. Pour des raisons familiales, ces situations sont complexes à gérer sur le plan professionnel et personnel. des organisations syndicales aux associations, en passant par nos concitoyens d'outre-mer, tous ont signalé différents manquements et retards quant à la mise en oeuvre de ce changement législatif dans les politiques de gestion des ressources humaines des différents ministères. Ainsi, le présent amendement vise à

relative à l'égalité réelle outre-mer. Deux ans après son entrée en vigueur, une circulaire du 1 mars 2017 est venue la préciser. Pourtant, les syndicats de fonctionnaires ultramarins n'ont de cesse de signaler les nombreux dysfonctionnements dans l'application du critère du centre des intérêts matériels et moraux comme priorité légale d'affectation. En effet, celui-ci ne s'appliquerait en réalité que depuis les mouvements de 2018. Qu'il s'agisse des difficultés rencontrées dans la constitution des dossiers ou de la non-rétroactivité de la loi par rapport aux dossiers déposés avant l'entrée en vigueur des dispositions, le dispositif pâtit incontestablement d'un manque de transparence et de clarté pour les fonctionnaires. C'est pourquoi nous demandons

je constate que c'est l'anniversaire de notre collègue, vice-président du Sénat, Thani Mohamed Soilihi, et je veux lui souhaiter un bon anniversaire.

Si le système de notation chiffrée était loin d'être parfait, le remplacement par l'entretien individuel dans la fonction publique territoriale et d'État a été très critiqué par les organisations syndicales, car l'individualisation de l'évaluation se fait au détriment des critères collectifs. La suppression de la notation aura des conséquences immédiates, par exemple sur l'attribution de la prime de service, si celle-ci est maintenue. L'article 12 du texte remplace donc la notation dans la fonction publique hospitalière, mais sans tenir compte de la situation de tension des personnels. Je vous renvoie à un débat que nous avons eu précédemment sur la précarité.

qu'il s'agisse des personnels souhaitant réfléchir à leur avenir et formuler des remarques sur le fonctionnement du service, ou des personnels encadrants, qui n'ont pas été accompagnés pour réaliser ces entretiens. Aujourd'hui, l'entretien individuel se résume à l'envoi aux agents, une semaine auparavant, de la fiche de poste et de la fiche d'entretien individuel, et à un échange avec l'encadrant n+1, durant vingt minutes, sur le bilan de l'année et sur les objectifs de l'année suivante.

professionnel annuel dans la fonction publique. Cette modalité d'évaluation, qui est déjà la norme dans les versants État et territorial, est attendue par les employeurs publics du versant hospitalier. Il est prévu que l'évaluation par entretien annuel entre en vigueur le 1 janvier 2021, et s'applique aux entretiens professionnels conduits au titre de l'année 2020.

Savoldelli. Sur l'expérimentation, je ne puis que regretter qu'elle n'ait pas été développée. Pourtant, Mme la rapporteur l'a dit, les employeurs et une très large part des organisations syndicales sont favorables, de manière

de loi du 11 janvier 1984 précitée est ainsi rédigé : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. de loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi modifié : « L'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct. » Enfin, l'article 76 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, non modifié, quant à lui, par le présent projet de loi, est ainsi rédigé : « L'appréciation, par l'autorité territoriale, de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à l'établissement d'un compte rendu » Il arrive cependant que cet entretien ne soit pas possible, en raison d'une situation de conflit,

il y aura de moins en moins de promotion interne. En réponse, la commission a prévu de calculer les ratios de promotion à partir du nombre non seulement de fonctionnaires, mais également d'agents en contrat à durée indéterminée. Cette disposition nous semble bien relever du domaine de la loi, car elle concerne la libre administration des collectivités territoriales.

Je serai bien sûr attentif, après avoir écouté M. le ministre de l'éducation nationale dans cet hémicycle, à son utilisation par le ministère de l'éducation nationale. Je ne reviendrai pas sur ce que j'ai entendu au sujet des relations entre

qui implique qu'un fonctionnaire ne soit pas affecté à un service relevant d'une carrière et d'une grille indiciaire moindre que celle qui correspond au corps dont il relève. Nous soumettons donc la possibilité pour un fonctionnaire d'exercer des fonctions ne relevant pas,

de la commission ? Nous comprenons très bien les motifs de cet amendement, notamment pour certains personnels de l'éducation nationale. Néanmoins, dans les faits, si elle devait être appliquée à l'ensemble de la fonction publique, une telle disposition interdirait toute forme de détachement. Le principe est justement que l'on puisse momentanément quitter son corps pour un autre et mener une double carrière. Une telle mesure créerait un frein brutal à la mobilité dans l'ensemble de la fonction publique, alors que les agents ont des attentes de plus en plus grandes en la matière. C'est la raison pour laquelle nous sommes défavorables

Les décrets fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois créent un parallèle entre niveau de responsabilité et taille de la collectivité. Par conséquent, les cadres de la fonction publique territoriale travaillant en zone rurale, dans des collectivités moins peuplées, sont pénalisés, car ils sont considérés comme assumant moins de responsabilités que les cadres des collectivités plus importantes en nombre d'habitants. Or les agents des collectivités rurales doivent avoir les mêmes chances d'évoluer dans leur carrière que les autres agents de la fonction publique territoriale. C'est ce que nous proposons d'assurer avec cet amendement. Quel est l'avis de Cet amendement vise les seuils démographiques dans la fonction publique territoriale. Il existe en effet plusieurs seuils fixés par la loi ou le décret pour la création des emplois fonctionnels, les recrutements directs, notamment de certains cadres d'emplois comme les administrateurs territoriaux, territoriaux, et la promotion interne. En mai dernier, notre collègue Patricia Morhet-Richaud a posé une question écrite sur ce sujet. Elle prenait l'exemple des attachés territoriaux, qui doivent avoir exercé dans une commune de plus de 10 000 habitants pendant au moins huit ans pour accéder au grade d'attaché hors classe. d'un vrai sujet, mais qu'il est difficile d'aborder par voie d'amendements. Il serait préférable que le Gouvernement s'engage dans une révision globale des seuils applicables à la fonction publique territoriale, en concertation avec les employeurs, mais également avec les représentants des différents cadres d'emplois. Enfin, je rappelle que la commission a déjà fait un pas en matière de promotion interne. Les quotas seront désormais calculés à partir du nombre total de fonctionnaires dans la collectivité, mais également en fonction du nombre d'agents en CDI. Comme j'aurais dû le faire pour l'amendement précédent, je demande le retrait, faute de quoi j'émettrais un avis défavorable. monsieur le ministre,

la nomination au tour extérieur des conseillers maîtres la procédure des examens de candidats, qui existe déjà pour la nomination au tour extérieur de conseillers référendaires. Quel est l'avis de

de la Cour des comptes. Aujourd'hui, ces rapporteurs peuvent être des magistrats ou des fonctionnaires appartenant aux corps recrutés par la voie de l'ÉNA ou des fonctionnaires ou des contractuels travaillant depuis plus de six ans à la Cour des comptes. Pour les auteurs amendement, les rapporteurs devraient désormais justifier de six ans d'ancienneté dans la fonction publique à l'intérieur ou à l'extérieur de la Cour des comptes. Nous comprenons la logique : attirer de nouvelles compétences au sein de la cour. Toutefois, cette disposition risque de désavantager les agents qui travaillent à la cour depuis de nombreuses années. Il semble donc difficile d'adopter cet amendement sans mettre en oeuvre un processus de concertation. Nous n'avons pu auditionner le Premier président de la Cour des comptes ; aussi, nous sollicitons l'avis tend à revoir la procédure de nomination des conseillers maîtres à la Cour des comptes. Aujourd'hui, deux tiers des nominations bénéficient aux conseillers référendaires, le reliquat étant partagé entre le tour extérieur et les membres des chambres régionales des comptes. Avec l'adoption de l'amendement, les conseillers référendaires seraient renforcés pour représenter trois quarts des nominations au grade de conseiller maître. L'objectif est de rajeunir ce dernier grade. Il s'agit toutefois d'une modification profonde de la Cour des comptes, qui nécessiterait une phase de concertation au sein même de l'institution. En outre, l'amendement a pour objet de renforcer les procédures du tour extérieur, en prévoyant un avis conforme d'une commission siégeant auprès du Premier président.

J'ajoute que nous ne souhaitons pas préempter les conclusions de la mission confiée à Frédéric Thiriez sur la gestion des carrières et les modalités de recrutement des hauts fonctionnaires.

Mme Éliane Assassi, sur l'article. J'interviens sur l'article 13 au nom de ma collègue Laurence Cohen, qui a dû s'absenter. En 2010, le Gouvernement Sarkozy avait introduit dans la fonction publique le versement d'une prime aux services ayant manifesté le plus d'« effort collectif » ou de « performance collective Le bilan n'est pas glorieux ! En effet, depuis 2010, seulement une dizaine de services de l'État et certaines collectivités ont mis en place une prime d'intéressement à la performance collective des services. L'article 13 du projet de loi reprend cet intéressement collectif et l'étend à la fonction publique hospitalière, où il était resté inappliqué. La prime d'intéressement collectif est versée aux agents en fonction non pas des résultats de l'agent, mais des résultats du service dans son ensemble. À l'hôpital, les réductions de moyens et les suppressions de postes ont largement dégradé les conditions de prise en charge des patientes et des patients, comme nous le dénonçons régulièrement. En instaurant un intéressement collectif des agents titulaires et contractuels de la fonction publique hospitalière lié à la qualité du service rendu, les agents, qui sont dépendants des budgets votés par les parlementaires, vont donc être doublement pénalisés une dégradation de l'offre de soins dont ils souffrent et qu'ils dénoncent, d'un côté, et, de l'autre, ne percevront aucune prime liée à la qualité du service rendu, pour des raisons indépendantes de leur volonté. Cela montre toute l'hypocrisie des critères de mesures de la performance qualitative du service rendu ! Ces techniques de direction, importées du secteur privé, ne sont pas applicables au secteur public, dont les caractéristiques propres de mission d'intérêt général sont trop éloignées

devient maintenant la norme du service rendu ... Vous ne dites pas la vérité aux agents ; chacun jugera ! Pour ce qui nous concerne, cet article est à l'antipode des propositions que nous portons pour améliorer la fonction publique hospitalière.

des agents contractuels. Or, malgré des dispositions améliorées dans ce projet de loi, la prise en compte des qualités professionnelles de l'agent reste facultative. Ainsi, il apparaît nécessaire d'imposer la prise en compte du mérite en liant la rémunération de l'agent à ses résultats professionnels. Quel est Quel est l'avis de la commission ?

Comme le souligne l'étude d'impact adjointe au projet de loi, la prime d'intéressement prévue dans l'article 78-1 de la loi du 9 janvier 1986 relative à la fonction publique hospitalière « n'a n'a pas pu être mise en oeuvre par les établissements en l'absence de textes réglementaires d'application tenant à la difficulté de déterminer des critères homogènes d'attribution de l'intéressement pour les différents types de service ». Sans rappeler l'intégralité des faits déjà largement relatés lors de l'examen du projet de loi « santé », ni le contexte social actuel dans nos hôpitaux, qui se caractérise par la mise en grève de quatre-vingt-dix services d'urgence, nous nous félicitons que les dispositions nécessaires aient été introduites pour rendre l'article 78-1 opérationnel et faire ainsi émerger une forme d'intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière, au moment où la revalorisation du travail de ces agents est essentielle. Certaines modifications ont été introduites en commission des lois, notamment l'obligation de saisine préalable du comité social d'établissement, le CSE, par analogie avec la procédure prévue pour la prime d'intéressement collectif dans la fonction publique territoriale. Nous nous interrogeons simplement sur la nécessité de cette formalité, dès lors qu'elle n'avait pas été prévue dans le texte initial et que l'avis du CSE est non contraignant. N'y a-t-il pas là un risque d'alourdir inutilement cette procédure et de retarder la décision d'attribution de cette prime ?

La disposition en question tend à soumettre au comité social d'établissement la mise en place d'une prime d'intéressement collectif dans la fonction publique hospitalière. Cette consultation existe déjà dans la fonction publique d'État et la fonction publique territoriale. Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable.

? Je suis convaincu que ma collègue Nathalie Delattre ne m'en voudra pas de retirer cet amendement

à redonner du sens aux missions des agents territoriaux, en cessant d'appeler dans le même temps à la reconnaissance de leur mérite et à la suppression de leur poste dans une logique d'économies budgétaires de bout de chandelle ! Quel est

des résultats individuels. En outre, nous avons donné plus de souplesse aux zones les plus enclavées pour leur permettre de recruter des agents à fort potentiel. Enfin, je rappelle que l'article 13 prévoit également le maintien des primes pendant les congés de maternité et de paternité, ce qui nous semble constituer un droit supplémentaire pour les agents. Par conséquent l'avis de

Une mesure en ce sens serait susceptible d'emporter des effets difficilement mesurables, tels qu'un accroissement des inégalités salariales y compris au sein d'une même collectivité, ou encore des freins à la mobilité

Par conséquent, il reprend sur ce point la rédaction adoptée par la commission. Il reprend également, dans ce nouvel article, la disposition proposée par la commission de maintenir le régime indemnitaire des agents territoriaux en cas de congé de maternité, disposition qui figurait initialement à l'article 32 du présent projet de loi, mais qui trouverait aisément sa place dans cet article 13 . Quel est l'avis de la commission ? Nous avons trouvé un terrain d'entente avec le Gouvernement concernant la reconnaissance des résultats du service dans le régime indemnitaire tenant Elle constitue une grande avancée pour les collectivités, notamment pour mieux valoriser les agents qui assurent des missions d'exécution. La commission a également proposé que les collectivités territoriales rencontrant des difficultés particulières de recrutement puissent augmenter le montant de leurs primes, le cas échéant

qui doivent parfois venir d'autres régions, elles-mêmes éloignées du territoire de ces collectivités, au point qu'elles n'arrivent pas à recruter. Si nous étions sur un marché- c'est d'ailleurs ce que font les entreprises de ces territoires enclavés -, nous pourrions compenser l'effort

qui a davantage les moyens d'assurer ces mouvements de fonctionnaires. Par conséquent, quand cela est réellement justifié, c'est-à-dire les collectivités en cause ou leurs établissements publics rencontrent des difficultés particulières de recrutement, on devrait pouvoir recruter ces agents en leur offrant un régime indemnitaire convenable.

que l'État puisse intervenir dans le processus, à un moment ou à un autre, pour éviter des excès, par exemple, des justifications infondées. De cela, nous pourrions discuter. En revanche, sur le principe de la facilitation du recrutement de cadres de haut niveau dans les collectivités relevant de territoires enclavés ou éloignés, je crois qu'il nous faut absolument faire mouvement.

À l'occasion du rendez-vous salarial annuel que je tiendrai le 2 juillet avec les organisations syndicales, la question du Rifseep sera abordée, et nous chercherons, au travers de ce dispositif, à apporter des réponses à cette problématique. Toujours en matière de Rifseep, je réitère l'engagement- ou l'annonce, je ne sais quel terme employer -fait à l'occasion de la discussion générale. J'ai demandé à la direction générale des collectivités, ainsi qu'à la direction générale de l'administration et de la fonction publique, de préparer un projet de décret permettant de délier les calendriers de mise en oeuvre du Rifseep sur les cadres d'emploi de la fonction publique territoriale. Aujourd'hui, le principe d'homologie et celui de parité- mais surtout celui d'homologie -fait que les collectivités ne peuvent facilement déployer le Rifseep, notamment sur la filière technique, tant que l'État n'a pas fait son travail de déploiement du Rifseep sur les corps d'emplois techniques qui relèvent de sa compétence. La principale justification à cette liaison de calendriers tient au principe de parité et de plafonnement du régime indemnitaire des cadres d'emplois de la fonction publique territoriale par rapport aux cadres d'emplois en homologie dans l'État. J'ai demandé que soit préparé un projet de décret. Il s'agit de délier ce calendrier, dans le respect du principe de parité, quitte à envisager des dispositifs d'ajustement pour faire en sorte que ce plafonnement- puisque c'est à cela que l'on aboutit -du régime indemnitaire des cadres d'emplois de la fonction

et de la liberté d'action aux collectivités territoriales pour déployer le Rifseep. Nous travaillerons par ailleurs, à partir du 2 juillet, sur les critères mêmes du Rifseep pour le rendre plus attractif. Cela n'épuisera pas tous les sujets, mais je tenais à le signaler à votre assemblée.

M. Canevet propose de supprimer cette obligation. Je n'y suis pas favorable, pour deux raisons : tout d'abord, il convient d'encourager les employeurs à valoriser le mérite de leurs agents ; ensuite, les collectivités territoriales peuvent déjà, en l'état du droit, fixer le niveau du CIA à 0 %.